Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et le site internet du Sénat, ainsi que sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun d'entre vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges

restaurera la confiance des Français et redonnera de la valeur au travail. Ces affirmations, monsieur le Premier ministre, ne relèvent-elles pas de la méthode Coué ? Comment affirmer que le niveau des retraites ne faiblira pas, alors qu'elles seront calculées sur la durée totale des carrières ? Que les pensions versées aux femmes seront meilleures, alors que celles-ci subissent toujours les effets des écarts de salaire et de carrières parfois hachées ? Comment assurer aujourd'hui une valeur du point, alors que vous exigez d'ores et déjà que le poids des retraites dans le PIB n'excède pas 14 %, comme c'est le cas aujourd'hui, et que la valeur du point servira évidemment de variable d'ajustement ? D'ailleurs, comment la valeur du point sera-t-elle pilotée, et par qui ? La question n'est pas neutre, si l'on se réfère à mes remarques précédentes. Le principe du départ à 62 ans semble préservé, mais avec l'épée de Damoclès inacceptable d'une décote pour celles et ceux qui décideront de partir avant 64 ans. Inacceptable pour ceux qui exercent les métiers les plus contraignants et qui ont commencé à travailler tôt, dont le niveau de pension est plus faible et qui ne pourront se permettre le principe d'une baisse de leurs revenus. Inacceptable pour ceux, nombreux, qui à 62 ans déjà sont bannis du monde du travail. Alors, monsieur le Premier ministre, vous avancerez certainement des arguments tels que l'amélioration des retraites pour les plus modestes et certaines professions, comme les agriculteurs. Mais, au vu de toutes les incertitudes que je viens d'évoquer, même ces bonnes intentions peuvent être soumises à caution. En clair, vous allez nous proposer de passer d'un système qui n'est certes pas parfait

Les recommandations de Jean-Paul Delevoye sont, vous le savez, le fruit d'une très longue concertation, à la fois citoyenne et avec les partenaires sociaux ; la qualité de cette concertation a été soulignée par tous les acteurs ce matin.

Il ne m'appartient pas, à ce stade, de me prononcer sur telle ou telle proposition du haut-commissaire. Ce dont nous sommes convaincus aujourd'hui, c'est que, demain, le système universel sera plus juste, puisqu'il ouvrira les mêmes droits pour tous. L'équité et la justice sont les deux mots d'ordre de ce système universel des retraites : un euro cotisé vaudra la même chose pour les salariés, les fonctionnaires, les commerçants, les agriculteurs.

La deuxième étape de la concertation s'ouvre à présent, sur la base des propositions du haut-commissaire à la réforme des retraites ; elle se fera avec les parlementaires, les partenaires sociaux et avec nos concitoyens. La parole

Le Royaume-Uni a fait part de son inquiétude à la suite de l'arrestation d'une ressortissante irano-britannique. Les États-Unis et le Canada sont aussi concernés. Ces arrestations interviennent dans un contexte de montée des tensions entre Washington et Téhéran. Elles font suite au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, le 8 mai dernier. Le régime iranien met ainsi la pression sur les gouvernements concernés, afin de constituer une monnaie d'échange en cas de conflit. L'Europe a tenté de sauver l'accord sur le nucléaire en créant la plateforme d'échanges Instex, toujours inactive, ce qui laisse l'Iran subir de plein fouet les sanctions américaines. Faute d'autres solutions, Téhéran viole le traité et reprend sa marche vers l'arme nucléaire. Personne ne veut voir l'Iran se doter de la bombe nucléaire et, surtout, personne n'a intérêt au déclenchement d'un conflit. Pourtant, la guerre semble se rapprocher. L'Europe et la France sont prises en étau par cette montée des extrêmes. Nous ne pouvons que condamner le choix de Téhéran, sans pour autant approuver la décision du Président Trump. L'Iran ne doit plus être une menace pour la région. Deux réponses sont possibles : la militaire, qui serait l'option de tous les dangers, et la négociation, aujourd'hui à l'agonie. Monsieur le ministre, la France est désormais directement concernée par ces tensions. Beaucoup de faux pas ont été faits en restant immobile », disait Disraeli. Il nous faut donc agir ! Comment la France envisage-t-elle d'obtenir la libération de Fariba Adelkhah ? Comment éviter le pire ? La

dans le contexte du dépassement par l'Iran de deux limites posées par l'accord de Vienne, le niveau d'enrichissement de l'uranium et le stockage de celui-ci, notre priorité est claire il faut que l'Iran se remette sans délai en conformité avec ses engagements. C'est une question de principe s'agissant d'un accord signé, mais aussi, comme vous l'avez souligné, un enjeu de sécurité. Car le non-respect par l'Iran de ses obligations sûrement des tensions internationales déjà très fortes dans la région, où, vous le savez, la situation est grave. La France est pleinement mobilisée pour contribuer à la désescalade des tensions. ? Rappelons-nous pourquoi nous en sommes arrivés là : l'Iran a eu une mauvaise réaction à une mauvaise décision américaine, celle de se retirer du JCPoA et de prendre des sanctions

C'est ce pour quoi nous nous mobilisons, singulièrement le Président de la République, qui entretient des relations directes avec le Président Rohani et le Président Trump. C'est aussi le sens du communiqué publié par Mmes Merkel et May et le Président Macron le 14 juillet. Quant à la situation de Mme Fariba Adelkhah, nous la suivons de très près. Le Président de la République s'en est entretenu avec le Président Rohani. Nous avons demandé des informations nécessaires, nécessaires, l'accès consulaire et une libération rapide. Je constate que, aujourd'hui, nos demandes ne sont pas satisfaites. Il est donc indispensable et urgent que les autorités iraniennes se montrent transparentes sur ce dossier, comme sur tous les dossiers des ressortissants étrangers arrêtés en Iran.

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Dimanche dernier, jour de notre fête nationale, des supporters de l'équipe de football d'Algérie ont célébré la qualification de leur équipe pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations, ce qui a occasionné des actes de violence et de destruction dans Paris, Lyon, Marseille et bien d'autres villes. Ce ne sont pas moins de 282 personnes qui ont été interpellées cette nuit-là, dont 249 placées en garde à vue, selon les sources du ministère de l'intérieur. En revanche, la place Beauvau se refuse à révéler le nombre exact de voitures brûlées : cette omerta est incompréhensible ! Ces scènes Ces scènes de violence se sont répétées partout en France, scénario qui laisse présager le pire en cas de victoire ou de défaite de l'Algérie lors de la finale de demain. Monsieur le Premier ministre, il est choquant et révélateur de voir cette nuée de drapeaux algériens brandis par des Français issus de l'immigration, dont les parents ont délibérément fait le choix de la France comme nouvelle patrie. il est choquant d'assister à ce type de manifestations violentes, surtout le jour de notre fête nationale. Des violences que l'État donne l'impression d'accepter comme une fatalité et qu'il ne gère qu'au coup par coup. Les Français en ont assez. Il est temps de ramener la paix sociale dans notre pays en recréant une unité de valeurs républicaines, sans favoriser, comme c'est le cas aujourd'hui, les communautarismes de toutes sortes. Cette violence est révélatrice d'un problème plus profond, plus grave

Monsieur le Premier ministre, la politique de l'autruche n'a que trop duré ! Il faut conclure ! Quelles réponses concrètes le Gouvernement compte-t-il enfin apporter à ces dérives, à cette carence d'éducation civique, à ce mépris des valeurs qui font la France ?

La parole est à Mme Michèle Vullien, pour le groupe Union Centriste.

en marge de scènes de liesse et de joie bien compréhensibles, le fait d'amateurs de sport, des bandes organisées ont fait basculer un moment heureux et sympathique dans des excès qui heurtent et meurtrissent. Violences matérielles, violences symboliques, violences verbales et même violences physiques à l'encontre des forces de l'ordre : on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé ! Ces actes inqualifiables ont été largement relayés par les médias. Ainsi, j'ai vu à la télévision- sans donc être sur place -un magasin

Les incidents du soir prolongent des incidents de même nature survenus quelques jours auparavant et quelques mois plus tôt. Ils se renouvellent sans que nous soyons en mesure de faire régner l'ordre ni de rassurer la population, malgré la mobilisation d'un dispositif important, que vous venez, monsieur le secrétaire d'État, je m'interroge sur notre capacité à faire respecter les lois, à contenir ces déferlements de haine, à protéger, tout simplement, les personnes et les biens. À vouloir prendre trop de précautions, nous acceptons l'inacceptable, en ouvrant grand le champ à de dangereux amalgames ; et nous prenons de bien grands risques en poussant l'électorat modéré vers les extrêmes. vers les extrêmes. De manière globale, qu'avons-nous raté collectivement pour engendrer de tels déferlements de haine à l'égard de la France et de ses symboles ? Il faut conclure

Plusieurs rapports sénatoriaux ont souligné la nécessité d'une réforme systémique, l'impératif d'équilibre financier ne pouvant être la seule approche.

être engagé dès à présent ce débat national en posant le principe du passage progressif à un système par points [ ...], qui assurerait un lien plus clair entre cotisations et pensions, identifierait mieux les mécanismes de solidarité et serait un gage de clarté pour les jeunes générations, persuadées aujourd'hui anciens collègues étaient conscients qu'il fallait mettre fin aux additions de mesures paramétriques, qui ont transformé le système de retraite existant en un millefeuille indigeste. Une vraie réforme du système des retraites devrait être animée par les objectifs suivants : renforcer la solidarité intergénérationnelle en rendant le système intelligible pour tous ; mettre un terme aux iniquités entre actifs, notamment en fusionnant les 42 régimes pérenniser le système de manière durable en empêchant l'adjonction de réformes paramétriques. Répondre à ces objectifs, c'est répondre à l'engagement pris par le Président de la République devant les Français. Aujourd'hui, après deux ans de concertations, M. Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, a présenté son rapport aux partenaires sociaux, au Premier ministre et à vous-même,

je vous remercie pour votre question, qui me permet de compléter ma réponse à Mme Monique Lubin. Les préconisations du haut-commissaire constituent le socle de ce que devra être un système de retraite universel, mais il nous reste à définir les conditions de la transition vers ce système cible. Changer de système n'est jamais chose aisée, et il est indispensable que nous prenions le temps nécessaire, car il nous reste à arrêter les modalités pratiques du passage au nouveau régime ; il nous reste à rassurer et à apporter des garanties attendues par les Français sur ce qui touche leurs projets de vie les plus personnels et les plus longuement mûris il nous reste à prendre en compte de manière cohérente les exigences d'équilibre économique avant la bascule dans le nouveau système universel de retraite. Aujourd'hui, nous le savons, la retraite est un casse-tête, une injustice, parfois une angoisse. Un casse-tête quand il s'agit de comprendre ce à quoi on a droit.

qui n'ont pas confiance dans l'avenir. Le Président de la République s'est engagé à rendre notre système de retraite plus juste. Celui-ci doit rester généreux, tout en s'adaptant à une société où les gens ont plusieurs métiers et plusieurs statuts dans leur vie. Les retraités sont un pilier de notre modèle démocratique : ils font vivre la solidarité entre les générations et participent à la vie associative et citoyenne. Nous devons donc prendre le temps de préparer un système de retraite grâce auquel chacun puisse bien vivre sa retraite, avec sérénité et dans la justice. Une deuxième phase de concertation s'ouvre à présent, sur la base des préconisations du haut-commissaire à la réforme des retraites. Après ces concertations, le Gouvernement travaillera à l'écriture d'un projet de loi. C'est ce

je trouve totalement indécent que le licenciement de 1 900 personnes soit à peine relaté dans la presse nationale, quand on voit ce qui a occupé les flashs des chaînes d'information en continu ces derniers jours. Madame la ministre, les salariés craignent un plan de démantèlement caché qui suivrait le plan de restructuration. Le PDG de Conforama s'est engagé le 14 juillet, par voie de presse, à ne pas démanteler l'entreprise, qualifiant ce scénario de « fantasme intégral

de maintenir l'activité hexagonale, mais dont le produit de la vente ne sera pas alloué à la procédure ni aux salariés touchés. Par ailleurs, l'entreprise a perçu pour plus de 50 millions d'euros

Steinhoff. Au-delà de ces difficultés actionnariales, Conforama fait face, comme tous les acteurs de la distribution, à l'évolution très rapide des modes de consommation et à la concurrence croissante des acteurs de l'économie numérique, sur un marché du meuble qui s'est révélé particulièrement difficile en 2018. C'est dans ce contexte que la direction de Conforama a annoncé un plan de restructuration très important, comprenant notamment la fermeture de 32 magasins Conforama et de 10 magasins Maison Dépôt. Je comprends l'angoisse et la colère des salariés face à ces annonces. Bruno Le Maire et moi-même sommes très fermes : il est indispensable que le dialogue puisse avoir lieu, et que les représentants du personnel obtiennent rapidement les réponses attendues sur la stratégie du groupe.

C'est pourquoi j'appelle la direction comme les organisations syndicales à poursuivre le dialogue, qui doit être transparent et loyal. Bruno Le Maire et moi-même serons particulièrement attentifs aux conditions de mise en oeuvre de la restructuration engagée par le groupe, qui doit donner à l'entreprise toutes ses chances de rebondir.

Zineb Redouane, octogénaire, morte après avoir été atteinte au visage par une grenade lacrymogène alors qu'elle fermait ses volets. Geneviève Legay, militante d'Attac, 73 ans, blessée à la tête à la suite d'une charge de CRS. Près de 3 000 blessés parmi les « gilets jaunes », 94 gravement, des mutilés, des éborgnés ! Face à cela, quoi donc ? Des enquêtes de l'IGPN ne débouchant sur rien ! Face à cela, quoi encore ? Un Président de la République, le 7 mars, jugeant « inacceptables » les mots de « répression » et de « violences policières » dans un État de droit. Ce ne sont pas les mots qui sont inacceptables, mais les faits ! Or les faits sont là, incontestables. Dernière affaire en date, celle de Steve Maia Caniço. Dans la nuit du 21 au 22 juin, à Nantes, des policiers interviennent contre des jeunes célébrant la fête de la musique un peu trop tardivement. On a parlé de lancers de projectiles ; les vidéos disponibles n'en montrent aucun. À la suite d'une charge visiblement disproportionnée, 14 personnes sautent dans la Loire pour échapper aux coups et aux grenades lacrymogènes. Steve, lui, n'a pas été retrouvé. Des enquêtes ont été diligentées, des plaintes ont été déposées, le Défenseur des droits s'est autosaisi. La famille de Steve, elle, attend toujours des réponses. Ma question est simple, monsieur le secrétaire d'État : où est Steve ? Je répète : où est Steve ? La

qui se sont déroulés pendant le mouvement des « gilets jaunes ». Systématiquement, quand des personnes ont été blessées, il y a eu saisine de l'autorité judiciaire. Ces investigations sont en cours. On relève plus de 280 saisines de l'Inspection générale de la police nationale. Plus d'une centaine de dossiers ont été transmis au parquet

Une action de police a été menée. Je vous rappelle qu'une action judiciaire a été engagée. Un juge d'instruction est saisi. Les investigations sont en cours, et ce n'est pas moi, en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, qui répondrai à des questions portant sur des investigations judiciaires en cours. Je sais simplement qu'elles sont menées très rigoureusement très sérieusement, et que toute la vérité sera faite sur cette affaire. Où cette réponse n'est certes pas de nature à calmer les inquiétudes de la famille de Steve. Le 16 juin dernier, dans le cadre de la mal nommée promotion « gilets jaunes », vous avez décoré M. Grégoire Chassaing, commissaire divisionnaire à Nantes. Cinq jours plus tard, le 21 juin, si l'on en croit Mediapart c'est le même qui ordonnait de gazer les jeunes rassemblés près d'une berge de la Loire. Il faut conclure Votre police va mal, monsieur le secrétaire d'État, et notre pays avec elle

Cela se passe à Paris, mais aussi à Rennes, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, à Saint-Denis, à Toulouse, et ailleurs encore. Le 23 avril dernier, les maires de ces villes ont interpellé ensemble le Gouvernement pour réclamer le renforcement des dispositifs d'accueil des réfugiés. Bien sûr, les municipalités mettent en place, avec les associations, des mesures humanitaires d'urgence et des accueils de jour. Je veux d'ailleurs ici remercier et saluer l'ensemble des acteurs qui s'engagent à leurs côtés. Mais ces mesures d'urgence ne peuvent pallier l'absence de l'État. Elles n'exonèrent pas le Gouvernement de sa responsabilité de prendre en charge durablement et d'héberger tous ceux qui dorment à la rue ou dans des campements de fortune. Alors que, depuis des mois, la situation est dramatique dans le nord de Paris, autour de la porte de la Chapelle, votre silence et votre passivité sont inacceptables, car l'accueil et la mise à l'abri des réfugiés relèvent de la compétence du Gouvernement ! Alors, monsieur le secrétaire d'État, j'ai deux questions. Quand l'État assumera-t-il enfin pleinement ses responsabilités ? Quand votre Gouvernement mettra-t-il fin à une situation indigne de notre pays et des valeurs de la République ? La parole

inacceptables. Vous savez très bien que nous avons fait des efforts importants pour augmenter l'offre d'hébergement des demandeurs d'asile. Ce sont 107 000 places qui sont disponibles sur le plan national, après une augmentation extrêmement importante. Il y en a 22 000 à Paris.

le sénateur, que le Gouvernement est passif sur ce dossier. Il l'est ! Il est très actif, et il l'est aussi à l'égard de ses partenaires européens, pour essayer de refonder l'espace Schengen et d'améliorer ce dossier également du point de vue européen. Nous sommes dans l'action, nous ne sommes pas passifs, monsieur le sénateur

Cessez de considérer cette question de l'accueil des réfugiés uniquement avec l'oeil du ministère de l'intérieur ! Construisez une réponse adaptée avec les collectivités et les associations ! Enfin, soyez à la hauteur de la promesse humaniste qui était la vôtre !

a été de baisser la taxe affectée sur le foncier non bâti, afin de faire baisser les taxes que les agriculteurs paient à partir de leurs revenus et de leur donner ainsi plus de pouvoir d'achat. Je veux en tout cas réaffirmer que les chambres d'agriculture ont un rôle essentiel à jouer.

C'est une agglomération internationale qui implique deux cantons suisses et deux départements français. Je souhaite exprimer dans cet hémicycle la très forte inquiétude des élus du territoire genevois français à propos de la politique menée par le Conseil d'État du canton de Genève en matière de scolarisation des enfants des expatriés suisses domiciliés en France. Les autorités genevoises ont décidé de modifier unilatéralement le règlement sur l'enseignement primaire. Hormis quelques rares exceptions,

Le coût du report de charges pour les collectivités comme pour l'État se chiffre en dizaines de millions d'euros ! Je rappelle que les frontaliers travaillant à Genève paient leurs impôts sur le revenu à la source au canton de Genève, qui en conserve les deux tiers. Monsieur le ministre, je souhaite connaître les initiatives que le Gouvernement entend prendre pour protester au niveau diplomatique le plus élevé contre des décisions qui affectent la vie quotidienne des habitants et des élus de toute l'agglomération. La parole est à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, la question que vous soulevez fait partie intégrante des discussions que nous avons régulièrement avec les autorités suisses, qu'il s'agisse des autorités fédérales ou, surtout, des autorités cantonales. Il est évident que notre coopération transfrontalière ne peut pas être déséquilibrée, qu'elle doit être juste et qu'elle doit se faire au bénéfice des deux côtés de la frontière. Dès l'adoption du nouveau règlement relatif à l'enseignement primaire à Genève, nous avons saisi les autorités cantonales pour souligner les difficultés et les implications d'une telle décision sur les capacités d'accueil et de scolarisation des établissements français frontaliers. Cette problématique a fait l'objet d'échanges nourris lors de la dernière réunion de dialogue transfrontalier. Les autorités cantonales genevoises sont restées sur leur position. Nous avons envisagé toutes les mesures permettant d'atténuer l'impact de cette décision, telles que la possibilité pour les élèves déjà scolarisés de terminer leurs études

Nous respectons les accords bilatéraux qui nous lient avec la Suisse et ses cantons, mais ces accords ne doivent pas nous empêcher d'améliorer les situations auxquelles nous C'est le cas, en particulier, dans le domaine de la coopération sanitaire transfrontalière, puisque nous avons conclu un accord à la fin du mois de juin. C'est le cas, aussi, de notre détermination à faire en sorte que la Suisse adopte, le plus vite possible, une directive sur l'indemnisation du chômage qui permettrait que les frontaliers soient indemnisés par le pays dans lequel ils travaillent, et non plus dans celui où ils résident. Voilà les enjeux de nos discussions. La situation transfrontalière entre la France et la Suisse est bonne, mais je constate avec vous qu'elle peut s'améliorer.

protectionniste inspirée par un populisme anti-frontalier qui se développe de manière préoccupante du côté suisse de la frontière. Nous devons être très vigilants sur ce point. La construction d'une coopération transfrontalière ne peut pas souffrir de telles décisions, à l'instar de la fermeture des petites douanes la nuit.

Pour reprendre ses mots, il s'agit d'« assurer notre défense de l'espace et par l'espace », « y compris de manière active ». Avec ce nouveau commandement, nous actons une évolution de notre doctrine militaire et nous faisons du domaine spatial une priorité stratégique et un véritable enjeu de sécurité nationale. Notre groupe salue une telle démarche, puisqu'elle permettra de rassembler nos moyens spatiaux, qui sont, pour l'heure, disséminés entre nos armées. L'espace exoatmosphérique n'est plus seulement un bien commun au service du progrès technologique humain C'est devenu un espace de conflictualité entre les puissances qui disposent de satellites, un espace à la fois disputé et contesté. Un satellite détourné de sa trajectoire, perturbé ou espionné, constitue une véritable menace pour la sécurité et la défense nationale, car ce satellite peut compromettre le fonctionnement de nos sociétés et de nos opérations militaires. C'est bien grâce aux satellites que nos militaires opèrent sur les théâtres d'affrontement, pour leur communication comme pour leur géolocalisation. Cela impose de renforcer notre vigilance quant à la sécurité et à la résilience de nos satellites. Monsieur le ministre, comment ce commandement de l'espace assurera-t-il la consolidation de nos capacités spatiales ? La loi de programmation militaire pour les avait déjà acté un renforcement du budget de la défense, qui doit augmenter à hauteur de 3,6 milliards d'euros. De nouveaux moyens seront-ils dédiés au renouvellement de nos capacités satellitaires et à la mise en oeuvre de cette nouvelle politique spatiale militaire ?

la ministre des armées, qui est actuellement en déplacement. Vous décrivez fort justement dans votre question l'enjeu de sécurité nationale que représente l'espace pour notre pays. C'est à la fois un enjeu de compétition, mais aussi, comme vous l'avez dit, un enjeu potentiel de conflictualités. Face à cet enjeu et- je dirais même -à ces menaces, nous avons décidé de renforcer notre action. Notre autonomie stratégique dépend en effet de notre capacité à sécuriser nos moyens spatiaux. Comme vous l'avez rappelé dans votre question, cette préoccupation était au coeur de la loi de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, qui prévoit le renforcement de nos capacités nationales de surveillance de l'espace exoatmosphérique et de connaissance de la situation spatiale, par le biais, entre autres, du renouvellement de tous nos satellites militaires de renseignement. La nouvelle stratégie spatiale de défense décidée par le Président de la République permet d'aller encore plus loin. Il s'agit désormais d'étendre notre surveillance des activités en orbite et de disposer des capacités nécessaires pour protéger, si besoin activement, nos intérêts spatiaux. À la suite des annonces faites par le chef de l'État, le 13 juillet, à l'hôtel de Brienne, comme vous l'avez rappelé, le grand commandement de l'espace qui sera créé d'ici à septembre au sein de notre armée de l'air rassemblera immédiatement 230 spécialistes. Il sera progressivement développé, tout particulièrement à Toulouse, siège du Centre national d'études spatiales, d'où nous mènerons nos opérations spatiales militaires. Mme la ministre des armées détaillera ce projet à Lyon, le 25 juillet prochain. C'est au travers de cet effort que nous protégerons nos satellites et nos moyens d'action dans l'espace, de contrer d'éventuelles menaces, et que nous garantirons l'usage pacifique de l'espace, dans le cadre fixé par les traités internationaux, auxquels le Gouvernement est particulièrement attaché. La parole

2 359 milliards d'euros, voilà le montant de la dette publique française au premier trimestre ! Ce n'est plus une petite montagne de dettes, c'est un Everest de dettes

Ainsi, une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de chaque Français. Face à cet Everest de dette, quel choix faites-vous ? Vous augmentez encore les dépenses publiques ! de 4,6 milliards d'euros, pour un budget de 267,5 milliards d'euros, alors qu'il existe des économies à faire en revoyant le train de vie de l'État, en réduisant le périmètre de la fonction publique, en réformant l'AME, ou encore en réévaluant l'efficacité des politiques publiques. J'en viens à ma question

son montant réel ! Près de 100 % du PIB ! Si les taux d'intérêt augmentent, vous faites courir une véritable catastrophe financière à la France ! L'épée de Damoclès s'abattra alors sur les Français. En ne faisant pas d'économies, vous faites courir un risque réel au pays. Il reste deux mois pour revoir votre copie. Le Sénat vous proposera des économies. Écoutez le Sénat !

des fréquences devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Bercy peut apprécier, puisque la cession des fréquences devrait lui rapporter entre 3 et 5 milliards d'euros. vous êtes face à un choix : soit tirer le maximum de profits pour l'État, soit imposer aux opérateurs des investissements permettant de couvrir rapidement l'ensemble du territoire, même le plus éloigné. Pour ce faire, il convient de baisser les recettes. Selon le choix qui sera fait, les déserts numériques en France s'accentueront ou reculeront. L'État a-t-il la volonté, monsieur le ministre, de faire de l'aménagement du territoire une priorité ? Malgré un discours qui se veut rassurant, il semble que l'État ait aujourd'hui choisi de privilégier les recettes. En 2025, deux tiers de la population seraient couverts, qu'un tiers ne le serait pas ! La fracture numérique va encore se creuser. Il ne faut pas renouveler les erreurs du passé. Le déploiement de la 4G avait privilégié les villes. N'oublions pas nos territoires ruraux ! Avec une recette aussi élevée que celle que vous escomptez, l'histoire risque malheureusement de se répéter. Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à renoncer à ces recettes pour permettre aux opérateurs, au travers d'un cahier des charges très exigeant, d'investir et de consacrer ces sommes à la disparition rapide et totale dans notre pays de la fracture numérique, qui alimente la fracture territoriale

vous l'avez dit, le cahier des charges des enchères 5G vient d'être soumis à la consultation publique par l'Arcep. Il reprend d'ailleurs les grandes orientations qui avaient été données par le Gouvernement en avril dernier. Je veux vous assurer que les objectifs du Gouvernement en la matière sont exigeants. C'est pourquoi nous souhaitons, notamment, mettre l'accent sur le développement des usages professionnels, par le biais de services différenciés, y compris dans les zones rurales. La volonté du Gouvernement est en effet- vous avez bien soulevé le problème sur ce point -de trouver un équilibre entre rendement et couverture du territoire.

Nous avons en particulier demandé que 20 % à 25 % des sites équipés le soient dans les campagnes comme zones de déploiement prioritaire, et ce dès 2024. L'objectif en effet n'est pas que les opérateurs fassent toutes les villes au début et les zones rurales à la fin. Ce déploiement sera donc rapide. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit : il est important de rappeler que les fréquences radioélectriques font partie du patrimoine de l'État. Nous avons ainsi tiré toutes les leçons des procédures d'enchères de nos voisins, pour que ce patrimoine soit valorisé, sans toutefois, je le répète, mettre en danger la capacité des opérateurs à déployer rapidement cette technologie sur tout le territoire. Le Gouvernement est en train de mener une étude de valorisation de ces fréquences afin de déterminer le montant des redevances qui seront associées à ces nouvelles attributions. Nous saisirons la Commission des participations et des transferts, qui devrait rendre un avis à ce sujet vers la fin du mois de septembre

la lutte contre la fracture numérique sont une priorité depuis des années. Naturellement, on compte sur l'engagement total du Gouvernement.

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'énergie et au climat.

en Europe. En France, quatre ports figurent dans le top 50 des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer.

est à Mme la ministre. Il est un point que je n'ai pas mentionné, car on est en train de parler de la pollution au soufre du transport maritime, mais il faut que chacun ait en tête que, en termes d'émissions de CO2 à la tonne transportée, le transport maritime représente 10 fois moins

français et étrangers, y compris à l'intérieur de la France, puisque la taxe de séjour serait comprise entre 20 centimes d'euros et 4 euros par nuit et par passager.

pose deux difficultés. D'une part, elle a de fortes probabilités d'être inconstitutionnelle, puisqu'elle traite différemment des contribuables, alors que le niveau de pollution n'a pas de rapport avec l'objectif d'une taxe de séjour, qui est notamment le développement des infrastructures touristiques.

Lors de leur stationnement en port, les grands navires de croisière continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques, le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote et les particules fines. La réglementation internationale en vigueur, bien qu'elle exige l'utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation, reste très peu efficace en la matière. Le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de teneur en soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis quinze ans pour celui des voitures- des voitures- 0,1 % contre 0,001 % -et le carburant qui sera utilisé massivement à partir de 2021 contiendrait

que l'ensemble des voitures circulant en Europe. En France, quatre ports figurent dans le top 50 des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer. À ce propos,

ailleurs- c'est la chimiste qui vous parle -, lorsqu'ils se combinent avec l'oxygène de l'air et l'eau qui est présente dans l'air, cela donne de l'acide sulfurique. C'est pourquoi ils attaquent les voies respiratoires,

a conclu que les émissions maritimes sont responsables de 60 000 décès prématurés en Europe en un an. Je reprends les propos de ma collègue Samia Ghali : à Marseille où la qualité de l'air est particulièrement préoccupante,

En effet, nous assistons depuis les ordonnances de 2016, ratifiées ici en 2017, à un recul du champ d'application de l'évaluation environnementale automatique au profit d'un examen au cas par cas, ce qui constitue à notre sens une sérieuse

En confiant aux services des préfets la décision de l'examen au cas par cas, les prérogatives de l'autorité environnementale sont de fait réduites, ce qui ouvre la voie à une multiplication des situations de conflits d'intérêts. Au

du droit. La réponse apportée à cette situation problématique est donc très largement insuffisante, mais également dangereuse pour l'environnement. Rappelons tout de même que toute activité humaine a une incidence sur l'environnement, et que, par voie de conséquence, tout projet devrait faire l'objet d'une évaluation de l'autorité environnementale. La parole La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l'article. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour l'heure, l'autorité environnementale, définie par voie de décret, a pour mission d'évaluer les incidences sur l'environnement de divers projets. Son rôle est primordial puisqu'elle se donne pour objectif de faire de la prévention écologique à l'échelle départementale. Pourtant, ses prérogatives avaient déjà été réduites par la loi ÉLAN, car il lui était reproché d'être un frein au développement de nombreux projets locaux. Ainsi, et progressivement, c'est le préfet qui a eu la charge de délivrer au cas par cas des autorisations de développement, lesquelles auraient à l'origine

Somme toute, ces derniers seront souverains dans leurs décisions, tandis que l'autorité, qui dispose d'une véritable expertise, jouera au mieux un rôle de conseiller. Au pire, elle ne sera qu'une simple chambre d'enregistrement soumise à la toute-puissance de l'administration. Alors que l'exécutif se donnait pour mission de rétablir une répartition rationnelle des compétences entre le préfet et l'autorité environnementale, il réduit le rôle de cette

qui s'en trouverait entravée. Alors que la transition énergétique devrait gagner en vigueur, certains signaux envoyés par le Gouvernement sont particulièrement décourageants.

a fixé des critères permettant de déterminer si les conséquences environnementales présumées du projet justifient une évaluation environnementale. Déterminer si elle est nécessaire est donc une compétence majeure, lourde de conséquences potentielles. Par ailleurs, cet article s'applique non seulement aux énergies renouvelables, mais également à des installations d'élevage, à la construction de certains aérodromes, à des barrages, des défrichements ou des rejets en mer. Il revient déjà au préfet d'autoriser ou non un projet, en tenant compte des aspects économiques et sociaux. En lui confiant également la tâche de déterminer si une évaluation environnementale environnementale est nécessaire ou non, on lui demande d'assumer plusieurs rôles tout en maintenant une apparence d'impartialité dans chacun de ses rôles. De plus, cette disposition multiplie les autorités à consulter : une pour le cas par cas, une pour apprécier la qualité de l'évaluation environnementale et, dans certains cas, une troisième en cas de modification d'un projet existant, voire une quatrième lorsque le projet nécessite l'évolution d'un plan. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. La parole

? Ces deux amendements de suppression me donnent l'occasion de revenir sur la réforme de l'autorité environnementale prévue par le Gouvernement à l'article 4 et sur ce que nous avons fait en commission. Actuellement, les projets de travaux et d'ouvrages susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale pouvant être, en fonction de seuils, soit systématique, soit effectuée au cas par cas, sur décision de l'autorité environnementale,

dans une décision du 6 décembre 2017, le Conseil d'État a annulé les dispositions permettant aux préfets d'être à la fois l'autorité chargée de donner un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet et l'autorité compétente pour autoriser ce projet, considérant qu'elles plaçaient les préfets en situation de conflit d'intérêts. L'article 4 du projet de loi prévoit par conséquent de séparer la fonction d'autorité chargée de l'examen au cas par cas des projets, qui pourrait être laissée au préfet, de celle d'autorité chargée d'émettre un avis sur l'évaluation environnementale des projets, qui serait confiée aux MRAE, lesquelles bénéficient d'une autonomie par rapport au préfet. Toutefois, cette solution continue de poser problème, puisqu'elle permet à un préfet d'être à la fois celui qui décide si un projet doit faire ou non l'objet d'une évaluation environnementale

Loin de sécuriser les porteurs de projet, la solution retenue par le Gouvernement pourrait donc aboutir à une multiplication des recours. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que l'autorité chargée du cas par cas devra bénéficier d'une autonomie fonctionnelle par par rapport à l'autorité compétente pour autoriser le projet. Au demeurant, c'est mot pour mot ce qu'a indiqué le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi.

les situations de conflit d'intérêts. Supprimer l'article 4 reviendrait à devoir confier l'examen au cas par cas des projets aux MRAE, or celles-ci ne sont pas dimensionnées pour traiter un tel volume de dossiers supplémentaires, ce qui risquerait d'allonger les procédures pour les porteurs de

je rappelle que le Conseil d'État a validé la rédaction du projet de loi sans la notion d'autorité fonctionnelle. Le Gouvernement ne souhaite donc pas qu'elle soit réintroduite dans le texte.

renforcer l'autorité environnementale et la rendre indépendante des autres pouvoirs administratifs. Or ce n'est pas du tout ce qui est prévu. C'est vrai

Le Conseil d'État a considéré dans une décision du 8 décembre 2017 qu'une réglementation qui exempte d'évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à obligation environnementale au cas par cas n'est pas conforme au principe de non-régression de la protection de l'environnement s'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

d'une évaluation. Cela ne serait pas compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle tous les projets ayant une telle incidence, y compris lorsqu'ils sont de dimension réduite, doivent être soumis à évaluation environnementale. Par cet amendement, nous souhaitons permettre à l'autorité compétente chargée de l'instruction du dossier de saisir l'autorité environnementale lorsqu'un projet se situant en deçà des seuils est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou sur la santé humaine. La saisine serait ouverte au maître d'ouvrage. La sécurité juridique des projets serait renforcée, puisque l'absence de réponse de l'autorité environnementale vaudrait dispense de réaliser l'étude d'impact. ainsi une recommandation du groupe de travail présidé par Jacques Vernier, qui préconisait une « clause de rattrapage ». Encore une fois, l'article 4 du projet de loi, combiné à cette lacune, constitue

pour autoriser des projets de saisir l'autorité environnementale afin d'examiner s'il est nécessaire de soumettre ces projets à évaluation environnementale, même s'ils sont en deçà des seuils fixés par décret. Le droit actuel fixe des seuils pour déterminer les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. La possibilité de définir de tels seuils est expressément prévue par la directive de l'Union européenne concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Je rappelle également que des discussions ont déjà eu lieu sur cette question à l'occasion de l'examen du projet de loi ratifiant les ordonnances du 3 août 2016 relatives à l'évaluation environnementale des projets.

est à Mme la ministre. En l'état de la législation, toute illégalité entachant les plans ou programmes pris en application du code de l'environnement entraîne leur annulation, même pour un simple vice de procédure qui pourrait être régularisé. Or l'approbation de ces plans et programmes est le résultat d'une procédure longue, incluant une concertation de l'ensemble des acteurs concernés, notamment les collectivités, les usagers, les riverains, afin d'identifier des solutions consensuelles à des problématiques qui peuvent être complexes. et ces programmes incluent notamment les plans climat-air-énergie territoriaux, les schémas régionaux climat-air-énergie, les plans de prévention des risques naturels ou technologiques, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Le présent amendement vise à étendre à ces plans et à ces programmes figurant au code de l'environnement la faculté ouverte au juge administratif par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour certains documents d'urbanisme, lorsqu'il constate qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de l'un de ces actes est susceptible d'être régularisée, de surseoir à statuer pour permettre à l'autorité administrative d'y procéder, ce qui lui évite de prononcer une annulation. Une annulation peut parfois être très lourde de conséquences, par exemple dans le cas des plans de prévention des risques technologiques, car elle augmente alors les risques pour les populations riveraines. Il convient donc que les vices de procédure qui peuvent être régularisés puissent l'être avant de prononcer l'annulation du plan programme.

plans de prévention des risques technologiques, notamment pour le déploiement d'installations produisant de l'énergie renouvelable. Sans autre précision, cette mesure nous semble dangereuse, car trop faiblement encadrée. En effet, si son auteur prend l'exemple de l'implantation de panneaux photovoltaïques dans les zones de mesures foncières délimitées dans le règlement du PPRT, rien n'indique que seuls des projets de ce type pourront provoquer des dérogations au plan de prévention des risques technologiques. Rien ne permet non plus de garantir que ces dérogations n'entraîneront pas une aggravation du risque technologique, technologique, ce qui serait alors contre-performant. En outre, confier cette possibilité de dérogation à la seule appréciation du préfet nous semble octroyer un pouvoir trop discrétionnaire à celui-ci. Pour l'ensemble de ces raisons, et alors que nous soutenons bien évidemment la multiplication d'installations d'énergies renouvelables, nous demandons la suppression de cet article, qui ouvre, à nos yeux, la voie à une remise en cause des plans de prévention des risques technologiques.

Mais encore faut-il que ce soit possible et que les conditions de sécurité soient réunies. Actuellement, il faut modifier le règlement du PPRT pour pouvoir procéder à de telles implantations. Or, vous le savez, la procédure est particulièrement lourde.

en accroissant le nombre de personnes nouvelles présentes dans les zones d'effets accidentels. Je suis évidemment défavorable à cet amendement. Monsieur Sueur, je n'ai pas connaissance des amendements qui n'ont pas passé le filtre de l'article 45.

Nous devons saisir cette opportunité pour lever les freins à l'industrialisation d'une filière émergente prometteuse dont les coûts baissent. Le prix était de 200 euros le mégawattheure lors de l'appel d'offres lancé en 2011, et les professionnels projettent un prix d'environ 50 euros le mégawattheure en 2025. Le rythme des appels d'offres doit s'accélérer si l'on veut réduire de moitié la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici à 2035 et assurer notre sécurité d'approvisionnement. Il faut aller plus loin et soutenir cette filière face à la massification du contentieux des énergies marines, qui nous fait prendre un retard considérable. Nous ne contestons pas, bien entendu, le droit au recours effectif, qui est un droit fondamental. Toutefois, la multiplication des recours ne doit pas aboutir à tuer les filières d'énergies renouvelables émergentes. Certes, des progrès ont été accomplis récemment en matière de traitement de ce contentieux, avec l'adoption du décret du 8 janvier 2016, lequel, en confiant la compétence des recours contre les énergies marines à la cour administrative d'appel de Nantes, a permis d'accroître la spécialisation de cette juridiction.

Nous avons en effet considéré qu'il existait déjà une procédure dérogatoire au droit commun : depuis 2016, le contentieux relatif aux énergies renouvelables en mer n'est pas porté devant les tribunaux administratifs, mais directement devant la cour administrative d'appel de Nantes, spécialisée

du Gouvernement ? Attribuer au Conseil d'État une compétence directe pour les projets d'énergie renouvelable en mer permettrait de réduire de douze mois en moyenne la durée des contentieux. Le lauréat d'un appel d'offres bénéficierait ainsi d'une meilleure visibilité sur le planning de développement du projet et pourrait engager plus rapidement et au meilleur coût la fabrication des composants, puis la construction de l'installation. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

sur l'article. Le dispositif des certificats d'économies d'énergie est un outil essentiel pour promouvoir et accompagner les économies d'énergie, avec le CITE, l'éco-prêt à taux zéro, les aides de l'ANAH

Grâce aux CEE, les économies d'énergie sont importantes. Elles ont lieu, pour 70 % d'entre elles, dans le bâtiment résidentiel. En 2018, 400 000 travaux d'isolation et 110 000 changements de chaudière ont pu être effectués grâce à ces certificats

ils considèrent que les démarches à accomplir sont très complexes. Par ailleurs, il m'est indiqué que le montant de l'aide n'est pas toujours adapté aux travaux. Soit il n'est pas assez incitatif,

des certificats d'économies d'énergie puisse rester efficace en matière de maîtrise des consommations. Il reste enfin à réagir face à l'augmentation des fraudes aux certificats d'économies d'énergie. Les dispositions de cet article me semblent particulièrement utiles et nécessaires pour

manque d'effectifs et n'ont conduit qu'à une cinquantaine de sanctions depuis 2015. Par ailleurs, un démarchage souvent agressif s'est développé au sein des entreprises réalisant les travaux, ce qui a conduit à rendre le dispositif relativement opaque.

un objectif global, mais aussi un chiffre pour les CEE normaux, un autre pour les CEE précarité, la fixation d'un taux de cotisation de chèque énergie et des franchises pour les petits fournisseurs. Le niveau

Afin de fixer les objectifs d'économies d'énergie à réaliser pour chaque période du certificat d'économies d'énergie, l'Ademe réalise des études évaluant les gisements d'économies accessibles. Pour les années à venir, nous pensons qu'il est important que cette évaluation donne une perspective de long terme, à dix ans, et permette une anticipation suffisante, en étant publiée au moins un an avant le début de la période d'obligation de ce certificat.

Par ailleurs, il apparaît opportun de supprimer la disposition qui bride les dates de la quatrième période d'obligation, afin de pouvoir prolonger celle-ci d'une année, jusqu'en 2021, comme cela est instamment demandé par la quasi-totalité des parties prenantes au dispositif.

l'objectif visé supposerait de connaître très précisément, pour les dix prochaines années, les coûts de l'énergie, ceux des travaux et des équipements, ou encore la propension des ménages et des entreprises à engager des travaux compte tenu des incitations financières proposées. Or cela dépend aussi du contexte économique.

aux demandes de CEE devront être effectués par des organismes d'inspection accrédités ; des vérifications supplémentaires sur trois ans d'opérations devront être faites après toute première sanction ; tous les acteurs auront l'obligation de signaler tout manquement aux règles de certification aux organismes qui les délivrent, qui devront à leur tour les examiner sans délai et en tirer les conséquences en matière de suspension ou de retrait de la certification.

et les organismes de certification, qui délivrent les certifications et prévoient déjà des contrôles pour vérifier la conformité des travaux aux règles de l'art. Ce sont non pas les premiers, mais les seconds qui peuvent conditionner l'octroi d'une qualification à telle ou telle condition. aller dans le sens souhaité par l'amendement, nous pourrions toutefois prévoir un pourcentage minimal de contrôles sur site devant être réalisés par l'organisme d'inspection.

correspondent à ce que les professionnels participant aux opérations « coups de pouce chauffage » ou « coup de pouce isolation » s'engagent déjà à faire en signant la charte de ces dispositifs. On cale donc le plancher sur les meilleures pratiques actuelles, ce qui est à la fois ambitieux et réaliste.

Le Gouvernement a engagé des travaux avec les parties prenantes afin de renforcer le dispositif de qualification RGE, notamment en matière d'audit périodique.

l'avis du Gouvernement ? Je comprends votre souhait d'améliorer les contrôles sur site pour les opérations d'économies d'énergie, mais il me semble important de moduler le taux de contrôles en fonction de la sensibilité des travaux et des problématiques détectées.

Outre les garanties apportées par l'accréditation, il convient de souligner que l'élaboration de rapports de contrôle biaisés constituerait une infraction pénale particulièrement grave pour l'organisme accrédité. Par ailleurs, la notion de lien capitalistique, juridique ou économique me semble vague pour constituer une interdiction de recourir à certains organismes. En outre, cette disposition pourrait manifestement être sanctionnée par le Conseil constitutionnel comme une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce ou de l'industrie.

aux seuls demandeurs, et non aux obligés qui achètent des CEE déjà délivrés de bonne foi. Cette précision permettra de traiter le vide juridique relatif à la question de la responsabilité du dernier détenteur sur la qualité d'un CEE, levant le risque juridique quant à

Madame la ministre, voyez-vous cet intérêt ?

Moga vise à mettre en oeuvre des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités locales financés par les obligés du dispositif CEE. Ces programmes permettraient notamment de financer l'ambition du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie « Encourager une rénovation une rénovation massive des bâtiments publics de l'État et des collectivités en mobilisant 4,8 milliards d'euros ». Ils pourraient être portés par un organisme public ou parapublic, finançant les projets de rénovation énergétique des collectivités locales les plus pertinents. Quel

au travers d'une plateforme permettant la cartographie, le ciblage, la standardisation d'opérations de rénovation énergétique des bâtiments éducatifs, avec une application en région Hauts-de-France. Le programme Énergie Sprong France a pour objectif un accompagnement de l'écosystème à la création et au développement d'un marché de la rénovation de très haute performance, notamment dans le secteur des bâtiments éducatifs, Le programme Actée a pour objectif de développer les projets d'efficacité énergétique des bâtiments publics et d'accompagner les collectivités. Elles peuvent également obtenir des CEE pour les travaux qu'elles réalisent sur leur patrimoine, ce qui peut représenter une contribution significative. Divers dispositifs de l'Ademe existent également, comme le conseil en énergie partagé. Enfin, 500 millions d'euros de dotation de soutien à l'investissement local sont mobilisés au sein du grand plan d'investissement pour cofinancer la rénovation thermique des bâtiments publics. J'ajoute que près de 2 milliards d'euros de prêts AmBRE sont mobilisables à la Caisse des dépôts et consignations, le taux de recours à ces prêts par les collectivités étant malheureusement aujourd'hui très faible.

car les principes généraux sont déjà clairement fixés dans la loi. En revanche, ce référentiel serait susceptible de devenir un outil supplémentaire pour les opérateurs de mauvaise foi, qui pourraient s'appuyer sur ce qu'il dit,

présenter l'amendement n° 10 rectifié. Il s'agit d'un amendement de notre collègue Jean-François Longeot. Les certificats d'économies d'énergie reposent sur une obligation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie. Les obligés devant promouvoir l'efficacité énergétique auprès de leurs clients, un marché des contrats a vu le jour. Ce marché s'appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d'économies d'énergie et donc de bénéficier de CEE. Ces bénéficier de CEE. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur en ne l'informant pas de l'existence d'un service public fournissant une information neutre. Cet amendement s'inscrit dans une optique de défense de l'accès à l'information du consommateur à l'établissement d'une convention entre la structure mettant en oeuvre le service public sur le territoire et les professionnels. Ces derniers devront systématiquement informer les consommateurs de l'existence du service public. La parole

le SPPEH. Il vise notamment à ce que les professionnels du secteur établissent une convention avec la structure mettant en oeuvre le service public sur leur territoire et informent systématiquement les consommateurs de l'existence de ce service public de la performance énergétique. Le consommateur aura ainsi les moyens de s'assurer de l'efficacité des travaux proposés. La parole est à M. il a été dit précédemment, la fraude aux certificats d'énergie, dont nous avions d'ailleurs dénoncé le potentiel spéculatif et les dérives frauduleuses, se répercute sur l'ensemble des ménages. En effet, le coût de ce dispositif, évalué entre 3 et 4 milliards d'euros, est financé sur leur facture énergétique. Pis, selon la Commission de régulation de l'énergie, l'augmentation des tarifs de l'électricité en août, après une augmentation de plus de 5 % début juin, sera en grande partie imputable aux certificats d'économies d'énergie. d'énergie. Dans sa délibération du 25 juin dernier, elle souligne : « Alors même que leurs bénéfices réels sont contestés, en l'absence d'évaluation approfondie du dispositif, et que des abus ou des fraudes sont régulièrement constatés, la hausse du coût des CEE explique la hausse de 1,23 % Si nous n'avons pas de chiffres précis, la fraude aux CEE peut être évaluée à plusieurs millions d'euros. C'est la raison pour laquelle nous avons repris cet amendement, proposé par Amorce, qui a pour objet de renforcer l'information du consommateur et le contrôle des professionnels

ou très vaguement, ce mécanisme et que de nombreuses arnaques ont été évoquées concernant des particuliers qui pensaient dépenser 1 euro et qui, finalement, devront payer plusieurs milliers d'euros, sans toucher les primes annoncées par l'entreprise. Comme le souligne Tracfin dans son rapport, la chasse aux CEE fait l'objet de campagnes de promotions massives auprès du grand public par mailing ou spots radiotélévisés de la part de sociétés fraudeuses. Tel est le sens de cet amendement, qui ne nous semble satisfait ni par le texte ni par le droit en vigueur. La

Le dispositif proposé pose cependant de nombreuses difficultés, comme je l'ai déjà dit en commission. En pratique, il existe aujourd'hui très peu de plateformes territoriales de la rénovation énergétique. À défaut, le texte renverrait la compétence aux EPCI

Il faut donc bien mesurer ce que vous proposez ! Enfin, quel serait le contenu de cette convention ? Quels engagements seraient pris et qui devrait les contrôler ? Il me semble que le dispositif de contrôle prévu à l'article 5, qui a été considérablement renforcé à l'Assemblée nationale que nous avons encore conforté, sera bien plus opérationnel, avec des obligations claires- contrôle préalable, vérifications supplémentaires en cas de première sanction -et des organismes pour les contrôler : organismes d'inspection accrédités et pôle national des CEE. Quant au service public de la performance énergétique de l'habitat, il s'agit effectivement d'un outil essentiel, mais qui tarde à se concrétiser dans tous les territoires. C'est avant tout une question de moyens, sur laquelle nous pourrons bien sûr revenir en loi de finances. La commission a émis un avis défavorable sur ces cinq amendements

mais également la réalisation de contrats d'entretien, l'installation de systèmes de récupération de chaleur, l'installation d'ampoules LED avec détecteur de présence dans des bâtiments tertiaires, les moteurs à variateur de vitesse, les dispositifs d'affichage de consommation ou encore les bornes de gonflage des pneumatiques. J'invite donc

avait sur la table environ 80 millions d'euros- madame la ministre, vous trouverez peut-être dans les archives trace de cette discussion -, financés notamment par la recette

Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service permettant de bénéficier de certificats d'économies d'énergie, au titre de l'article L. 221-7 du code de l'énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie

Le scrutin est ouvert.

en faveur des travaux réalisés dans les logements classés en catégories F et G. Dès lors que le résidentiel représente la principale source de consommation d'énergie primaire

Ces incitations bonifiées permettent de réduire très fortement le reste à charge des ménages, quel que soit le classement énergétique de leur logement, en particulier pour les ménages aux revenus les plus faibles,

de la discussion générale, des chercheurs suisses ont récemment mis en évidence que 900 millions d'hectares de canopée, en plus des 2,8 milliards d'hectares existants, permettraient d'absorber 205 des 300 gigatonnes de carbone émises dans l'atmosphère depuis le début du XIX siècle. C'est dire la puissance du levier de En France, la forêt représente 17 millions d'hectares et capte déjà 130 millions de tonnes de CO2 par an, soit 30 % des émissions. Par ailleurs, on constate que les fournisseurs d'énergie et les obligés accusent collectivement un retard de 40 % sur leurs obligations

Le prix des CEE est ainsi passé de 2 euros en 2016 à plus de 9 euros aujourd'hui. Le coût pour les consommateurs finals s'élève entre 100 et 150 euros par an et par ménage. Dans ce contexte, et afin d'accélérer la lutte contre les changements climatiques en optimisant les marges d'obligations non utilisées des CEE, cet amendement tend à proposer un nouvel outil, que nous avons appelé « certificat captation carbone », qui pourrait être ancré sur les CEE et qui fonctionnerait selon les mêmes dispositions, non en mégawattheures mais en tonnes équivalent carbone. offrirait la possibilité aux obligés de remplir leurs obligations liées à leurs émissions de gaz à effet de serre, en favorisant la captation de carbone supplémentaire par le financement de reboisement ou de restauration d'écosystèmes. Il permettrait ainsi aux forestiers, aux agriculteurs et aux collectivités locales de dynamiser la captation du carbone, en se réappropriant, par exemple, des friches industrielles, pour les renaturaliser, et en participant ainsi à la lutte contre l'artificialisation des sols. Je souligne pour finir tous les effets vertueux induits par cette disposition : augmentation de la séquestration de CO2 dans les sols, les végétaux et les matériaux en bois, lutte contre l'artificialisation des sols,

combien de fois avons-nous débattu, au sein de notre assemblée, des prestations pour les services environnementaux ? Ce serait une manière de reconnaître et de renforcer tous ces acteurs qui oeuvrent au quotidien dans la lutte contre le réchauffement climatique.

183. Outre le fait que le Gouvernement recourt de manière récurrente aux ordonnances, les auteurs de l'amendement estiment que le champ de l'habilitation prévue à cet article est beaucoup trop large pour être acceptable. en effet de transposer quatre directives et trois règlements européens, portant notamment sur un sujet de grande importance, celui de la transition énergétique, qui concerne concrètement, dans ses multiples dimensions, l'ensemble des citoyens et des territoires. À cela s'ajoute la transposition de la directive sur le marché intérieur de l'électricité, qui, eu égard aux enjeux qu'elle implique, mériterait à elle seule un projet de loi spécifique. L'examen de ces textes européens est en particulier nécessaire à deux titres. l'évaluation et la prise en compte des conséquences sociales de la mise en oeuvre des directives, en ce qui concerne l'efficacité énergétique et la performance énergétique des bâtiments, mériteraient des mesures nationales spécifiques d'accompagnement,

annoncé par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son programme, avec l'adoption d'ici à 2021 d'un plan complet visant à porter à 55 l'objectif de réduction des émissions d'ici à 2030, et avec la mise en place d'une véritable stratégie de l'investissement à destination de la transition écologique et énergétique. Nous avons besoin besoin d'évaluer ces directives à l'aune de ces nouveaux objectifs, d'autant que ce nouveau plan s'appuiera sur des analyses de l'impact environnemental, économique et social, analyses qui font d'ailleurs cruellement défaut aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain souhaite la suppression de l'article

commission ? Si le recours aux ordonnances n'est effectivement pas un procédé satisfaisant, la suppression de l'article ralentirait l'adoption des évolutions législatives qui doivent intervenir en application du paquet d'hiver, ce qui exposerait la France à une procédure en manquement, en cas de contrariété de sa législation avec le droit européen. En effet, l'entrée en vigueur de ces textes interviendra entre le printemps 2020 et le printemps 2021, un règlement étant d'ores et déjà entré en vigueur ; dès lors, le Parlement n'aurait que très peu de temps pour modifier la législation au regard de ces sept textes. Par ailleurs, dans son avis sur le projet de loi,

l'avis du Gouvernement ? Je comprends que le Parlement ne soit pas favorable au principe des ordonnances. Pour autant, les nouveaux textes européens sont extrêmement longs, techniques et détaillés, et ils ne laissent qu'une marge de manoeuvre très faible aux gouvernements pour leur transposition. Pour ces raisons, comme cela arrive fréquemment pour des textes transposant des directives, le recours à une ordonnance semble adapté, étant naturellement entendu que le Gouvernement associera les parties prenantes et M. le rapporteur,

membres de permettre aux ménages et aux collectivités de participer à une communauté d'énergie renouvelable, une CER, et d'établir un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, les amendement vise à intégrer dans le code de l'énergie les articles instituant les statuts des CER et des CEC, sans plus attendre,

activités, consolidant ainsi la transposition des directives au travers de l'article 6 A. Enfin, dans la directive 2018/2001, il est indiqué que les États membres doivent prévoir un cadre favorable

et 98 rectifié sont similaires. Les dispositions qu'ils tendent à insérer paraissent peu utiles au regard du texte existant. En premier lieu, les dispositions relatives aux communautés d'énergie renouvelable introduites par l'Assemblée nationale suffisent pour conférer

proposées par les amendements sur ce point sont donc de nature purement rédactionnelle. Par ailleurs, les modalités de fonctionnement que les amendements visent à instituer pour les CER, notamment, la coopération du gestionnaire du réseau pour les transferts ou l'absence de traitement discriminatoire, sont d'ores et déjà mentionnées.

dont elles sont issues. Le délai de transposition de cette directive étant fixé au 31 décembre 2020, il n'y a pas d'urgence à introduire en droit interne une notion dont on saisit encore mal les contours et les effets juridiques. En effet, alors que les CER ne visent qu'à produire, consommer, stocker ou vendre de l'électricité, les CEC ont d'autres missions, telles que la distribution de l'énergie ou la fourniture de services énergétiques. Cette différence de nature justifie que nous prenions davantage de temps pour transposer convenablement en droit interne les CEC, dont les implications juridiques sont plus nombreuses. Enfin, les modalités de fonctionnement des CER ne peuvent pas être appliquées telles quelles aux CEC, puisque la directive précitée prévoit des éléments spécifiques pour ces dernières,

En effet, tel que rédigé, l'article 6 A exclut cette possibilité, en contradiction avec les objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de à partir de sources renouvelables. L'article 2 de la directive laisse entendre que le secteur résidentiel est traité de manière différente des autres secteurs, puisque les termes « immeuble résidentiel » sont posés en alternative à l'expression « même bâtiment ». Par ailleurs, les considérants 66 et 67 de la même directive éclairent de manière précise l'intention du législateur européen, qui est de favoriser et non d'entraver le développement de l'autoconsommation collective, y compris dans l'objectif de réduire la consommation et de lutter contre la précarité énergétique. Il est donc nécessaire de revenir sur la limitation découlant de la rédaction de l'alinéa 15 de l'article 6 A. Quel est l'avis

En effet, l'article 21 de cette directive dispose que « les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d'énergies renouvelables situés dans le même bâtiment, y compris les immeubles résidentiels, aient le droit d'exercer collectivement [leurs] activités

du Gouvernement ? Comme l'a indiqué M. le rapporteur, la directive ENR de 2018 restreint sans ambiguïté l'autoconsommation collective à des opérations au sein d'un même bâtiment. amendement introduirait donc une disposition contraire à la directive européenne. Par ailleurs, l'article 6 A introduit en droit français une notion d'opération d'autoconsommation collective étendue, qui permet de répondre à l'objet de l'amendement. J'en demande donc le retrait.

électrique fine à une maille géographique d'un kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre. L'Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables, a modifié l'article L. 315-2 du code de l'énergie. Elle a cependant conservé une restriction au réseau basse tension des opérations d'autoconsommation collective, qui entraîne deux restrictions majeures. D'une part, cela signifie que les installations d'une taille supérieure à 250 kilowatts ne pourront pas entrer dans le champ de l'autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau haute tension. Le texte de l'arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3 mégawatts les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu'à 3 D'autre part, cela exclut des bâtiments dont l'importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C'est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les Ehpad, les petites et moyennes industries ou encore les supermarchés. ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de toitures importantes susceptibles d'accueillir une centrale de production solaire et de partager ainsi leurs électrons solaires. Cet amendement vise à revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s'inscrire sur le réseau de distribution d'électricité.

la définition des opérations d'autoconsommation collective pose trois difficultés. Tout d'abord, elle est susceptible d'engendrer un changement d'échelle, puisque l'on passerait de petites installations utilisant le réseau basse tension à des installations beaucoup plus puissantes, avec une transition sur le réseau moyenne tension.

et de solidarité nationale. J'étais d'ailleurs intervenu assez régulièrement sur ces questions, remettant même en cause un slogan qui avait fait florès à une époque dans un certain nombre de milieux favorables aux énergies renouvelables,

est à Mme la ministre. La loi Pacte a prévu que le ministre de l'énergie fixe par arrêté le périmètre des opérations d'autoconsommation collective et que cet arrêté soit signé après avis de la Commission de régulation de l'énergie. L'article 6 A prévoit d'aller plus loin en mettant en place un « avis conforme » de la CRE. Cette disposition, qui revient à transférer une mission additionnelle à la CRE, n'est pas conforme à ce qui a été voté dans la loi Pacte. Le présent amendement vise en conséquence à rétablir les dispositions votées. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 21 de la directive de 2018 sur les énergies renouvelables prévoit la possibilité, pour les États membres, de taxer l'autoconsommation. Les alinéas 20 prévoient que la CRE puisse établir des frais sur l'électricité autoconsommée dans un bâtiment, sans que la nécessité ou le besoin de nouveaux frais ait été démontré à ce stade. Dans la mesure où la directive laisse aux États membres le choix de mettre en place des frais sur les autoconsommateurs d'énergies renouvelables, que la nécessité de tels frais n'est pas démontrée et que la CRE n'a pas vocation à fixer des prélèvements, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 20 à 24. L'amendement n° 408, présenté

est à M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à clarifier le statut du producteur d'une opération d'autoconsommation collective et son lien avec les consommateurs finals, en précisant explicitement qu'il n'exerce pas une activité de fourniture au sens du code de l'énergie. l'énergie. La formulation de l'article L. 315-2 du code de l'énergie actuellement en vigueur peut laisser penser que le producteur participant à une opération d'autoconsommation collective est un fournisseur d'électricité et, par conséquent, que le régime juridique du fournisseur s'impose à lui, notamment en matière de contractualisation.

a indiqué que « l'autoconsommation collective permet d'approvisionner un consommateur en énergie sans passer par le cadre de la fourniture, et donc sans avoir à s'acquitter d'obligations prévues pour les fournisseurs ». Dès lors, il n'est pas souhaitable de modifier le code de l'énergie sur ce point. La commission a émis un avis défavorable

pour les communautés d'énergie renouvelable, conformément à ce qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Il semble prématuré d'instituer des garde-fous, alors que les initiatives d'autoconsommation collective peinent à voir le jour et que la directive 2018/2001 relative aux énergies renouvelables dispose en son article 22 que « les États membres prévoient un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d'énergie renouvelable À ce titre, les communautés d'énergie renouvelable doivent être soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes ainsi qu'à des frais d'accès au réseau reflétant les coûts. Elles doivent contribuer de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global des réseaux de distribution. Il est encore temps d'instaurer un cadre adapté aux projets d'énergies renouvelables portés par les acteurs du territoire.

de traiter ces communautés « d'une manière non discriminatoire » dans l'accès aux réseaux est consacrée par l'article 22 de la directive du 11 décembre 2018. Cette disposition pose également un problème au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, étant donné qu'elle conduirait à appliquer deux tarifs différents à des opérations d'autoconsommation identique dont la seule différence serait le statut juridique. L'avis est donc défavorable. Quel est du Gouvernement ? Je pense que cet amendement est satisfait. Des communautés énergétiques citoyennes peuvent, si elles le souhaitent, mettre en place une opération d'autoconsommation dite étendue. Dans ce cas, la communauté est la personne morale au sens du code de l'énergie. Dès lors, il ne semble pas nécessaire d'insérer l'ajout proposé par l'amendement, qui mélange le statut de communauté avec la réalisation d'opérations d'autoconsommation. Cela étant, je m'en remets à la sagesse du Sénat. La parole est

incitant au développement de ce mode de production et de consommation.

ou que sa participation à une communauté d'énergie renouvelable ou à une communauté énergétique citoyenne soit l'objet principal de son activité professionnelle ou commerciale. Une telle restriction est en contradiction avec l'ajout, opéré par la même commission, d'une définition légale du tiers-investissement dans

Ce tiers-investissement permet à une société de développer, financer et entretenir une installation de production renouvelable pour le compte d'un consommateur final autoconsommateur. Or, par l'alinéa 27 de l'article 6 A, il est interdit à cette activité de tiers-investissement de constituer une activité professionnelle ou commerciale principale. Il y a donc une contradiction manifeste entre ces deux propositions, qu'il convient de résoudre en supprimant les alinéas 26 et 27.

article modifie les dispositions relatives à l'autoconsommation et introduit la notion de « communautés d'énergie renouvelable », conformément à certaines dispositions du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens en l'état actuel, il ne comporte pas certains éléments permis par le droit européen et utiles à la régulation de l'autoconsommation, particulièrement pour ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, celles-ci ayant le droit d'être propriétaires de réseaux de distribution, ou de les établir, de les acheter ou de les louer et de les gérer de manière autonome. Il est étonnant que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale limite et encadre l'activité des membres des communautés énergétiques citoyennes, sans auparavant les définir. Je vous propose donc la suppression des deux alinéas encadrant cette activité, en laissant au décret d'application le soin de préciser l'activité des membres des communautés énergétiques citoyennes. La parole

vise à préciser explicitement que l'interdiction faite à une entreprise de tirer d'une opération d'autoconsommation une activité professionnelle ou commerciale à titre principal ne s'applique pas au tiers institué par le présent article.

409 visent à revenir sur le principe introduit en commission selon lequel, lorsqu'une entreprise participe à une opération d'autoconsommation, cette participation ne peut constituer son activité économique. Cette interdiction est issue de la directive du 11 décembre 2018, selon laquelle les activités exercées par des « autoconsommateurs d'énergie renouvelable » ou des « communautés d'énergie renouvelable » ne peuvent constituer une activité commerciale ou professionnelle à titre principal. ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, le considérant 44 de la directive du 5 juin 2019 indique que « les pouvoirs de décision au sein d'une communauté énergétique citoyenne devraient être limités aux membres ou actionnaires qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle L'interdiction faite aux entreprises de retirer une activité économique ou professionnelle à titre principal de leur participation aux opérations d'autoconsommation est donc largement étayée par le paquet d'hiver. C'est la raison pour laquelle la commission a transposé ces dispositions dans le code de l'énergie, afin de garantir que l'essor de l'autoconsommation demeure un mode de production d'énergie alternatif mobilisant des citoyens et des collectivités territoriales, et non une activité mercantile au premier chef. Cette interdiction n'a pas vocation à s'appliquer aux tiers gérants ou exploitant

j'ai presque l'impression que c'est un gros mot -et d'en être gestionnaires. Il s'agit de corriger une erreur de transposition de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est proposé de revenir sur cette interdiction faite aux communautés énergétiques locales, car elle entre en contradiction avec l'article 22 de la directive, qui prévoit explicitement cette faculté en mentionnant que ces « communautés d'énergie renouvelable ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations

224 rectifié et 410 visent à supprimer l'interdiction faite aux communautés d'énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes de détenir ou d'exploiter un réseau de distribution, largement confortée par la commission.

du Gouvernement ? Je m'étonne vraiment de ces amendements. La directive prévoit la faculté pour les États membres d'autoriser ou non les communautés énergétiques locales à détenir les réseaux. Il s'agit non d'une obligation, mais d'un choix de l'État. Le Gouvernement est convaincu de l'importance du réseau public, facteur de solidarité entre les territoires, notamment en faveur des territoires ruraux. Il est ainsi opposé à la possibilité pour des communautés énergétiques de posséder leur propre réseau. L'avis est donc défavorable

n° 46 rectifié. Cet amendement de Mme Estrosi Sassone vise à faciliter les projets d'autoconsommation collective portés par les organismes d'HLM disposant d'un fort potentiel de développement d'installations photovoltaïques sur leurs bâtiments.

d'habitations à loyer modéré de prendre part à des opérations d'autoconsommation collective sans créer une nouvelle personne morale.

autour de laquelle sont organisées ces opérations. C'est particulièrement regrettable, dans la mesure où les immeubles d'habitation de type HLM constituent un lieu favorable à la mise en place de ces opérations, eu égard à l'importance de la surface qu'ils occupent et de la population qu'ils hébergent. Dans ces conditions, la simplification proposée par les auteurs des amendements identiques est tout à fait utile.

le cas des HLM n'a pas besoin d'être conservée, puisque l'article 6 A, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, a introduit la notion d'opération d'autoconsommation collective dite étendue, qui permet de déroger à de stricts critères géographiques. D'autre part, le renvoi à un décret en Conseil d'État plutôt qu'à un décret simple semble plus protecteur sur le plan juridique, d'autant que les relations contractuelles entre les bailleurs et les locataires sont en jeu.

du Gouvernement ? Le Gouvernement est favorable au développement des opérations d'autoconsommation collective, qui peuvent être utiles et opportunes pour les bailleurs sociaux. Actuellement, rien n'empêche les bailleurs sociaux de devenir des personnes morales au sens du code de l'énergie

est à Mme la ministre. Actuellement, le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital de sociétés « dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité ». Toutefois, la notion de « territoires situés à proximité » pose des difficultés d'interprétation susceptibles d'affecter la sécurité juridique des prises de participation

c'est par l'intermédiaire d'une société dont l'objet consiste à investir dans les sociétés de production d'énergie renouvelable. Or l'article L. 2253-1 ne permet qu'une participation directe au capital de sociétés de production d'énergie renouvelable. Une intervention indirecte au travers d'une structure intermédiaire n'est donc pas possible possible en l'état. Cet amendement tend à lever un tel obstacle tout en définissant plusieurs limites. De plus, l'article L. 2253-1 ne porte que sur la prise de participation au capital. Or, outre la participation au capital, le financement des projets dans le secteur de la production des énergies renouvelables repose également sur l'octroi d'avances en compte courant émanant des actionnaires ou des associés de la société.

est très attendu par les territoires.

Mme la ministre.

nous considérons que l'intérêt général national commande de conserver la souveraineté sur la gestion de ces biens communs et de ces infrastructures stratégiques que sont nos barrages hydroélectriques. Car il s'agit bien d'un secteur stratégique, tant pour la production d'électricité renouvelable que pour la gestion des ressources en eau ! Je parle non pas de la propriété des barrages, qui demeurera évidemment

a pour objet de ne pas imposer une redevance, notamment lorsque la rentabilité de la concession ne s'améliorerait qu'à la marge. Une telle obligation pourrait être contre-productive ; elle ne va pas favoriser le développement de l'énergie hydraulique. Or l'objectif du présent dispositif est de permettre des augmentations de puissance hydro sur des concessions en cours sans obtenir en échange une prolongation. Pour augmenter la puissance, le concessionnaire doit investir. Afin qu'il puisse le faire, l'investissement doit être rentable. rentable. Si toute rentabilité donne lieu à une redevance de même montant, cela n'incitera pas le concessionnaire à investir, donc à atteindre l'objectif d'augmenter la production hydraulique. Il n'y a pas de lien absolu entre augmentation de puissance et équilibre économique. Une augmentation de puissance de 20 % n'aurait pas systématiquement pour effet une modification de 20 % de l'équilibre économique. Cet amendement vise à revenir sur l'une des modifications apportées en commission. Je le rappelle, la commission a cherché à consolider et à simplifier encore la possibilité offerte par l'article d'augmenter la puissance des installations hydroélectriques concédées sans remise en concurrence. En voulant limiter l'application de la redevance hydraulique, qui est notamment perçue par les collectivités, aux seules modifications substantielles de l'équilibre du contrat, on introduirait une contradiction avec le deuxième alinéa. Celui-ci prévoit que l'augmentation de puissance n'est possible que lorsqu'elle n'implique n'implique pas de modification substantielle du contrat lui-même. Par construction, elle ne peut donc pas conduire à modifier l'équilibre économique du contrat de manière substantielle. Si modification de l'équilibre économique il y a, il est logique qu'une redevance soit perçue pour rétablir l'équilibre économique du contrat et ne pas occasionner de surrémunération

du Gouvernement ? L'article 6 B ne permet de réaliser des augmentations de la puissance hydroélectrique que si les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concessions ne sont pas substantielles. Dès lors, il est impossible de prévoir qu'une redevance ne sera intégrée qu'en cas de modification substantielle sur le contrat, ce qui est par définition exclu du champ de l'article. J'invite donc les auteurs de cet amendement à le

L'article 6 B introduit un dispositif de « silence vaut accord » pour autoriser les augmentations de puissance des concessions hydroélectriques. Nous pensons qu'il serait préférable de le remplacer par une procédure de « silence vaut refus ». Il ne semble pas opportun de ne prévoir aucun accord explicite de l'État. de l'État. Dans la mesure où une telle augmentation nécessite en pratique une modification d'un contrat de concession, la procédure actuelle conduirait à des signatures tacites d'avenant à des contrats de concession. Aucun contrat ou engagement de l'État ne fait actuellement l'objet d'une signature tacite. Cette disposition créerait un précédent pour l'État dans ses relations contractuelles.

dans le développement de centrales solaires. Elle relève du classement des plans locaux d'urbanisme, et leur changement d'usage est déjà strictement encadré. Il n'y a donc pas lieu de restreindre ainsi les implantations en bord de réseau routier. Ces dernières pourront s'effectuer dans les mêmes conditions et avec les mêmes contraintes que sur le reste du territoire.

égard, je souhaite apporter une précision par rapport au débat que nous avons eu en commission. L'utilisation de terres agricoles n'est pas proscrite dans le développement de centrales solaires ; elle est simplement encadrée. Par exemple, un projet photovoltaïque doit permettre l'exercice d'une activité agricole significative sur le terrain d'implantation, mais la notion d'« activité agricole significative » n'est pas définie et est sujette à incertitudes. Il y a donc bel et bien un risque que les perspectives financières liées à un tel projet conduisent à une

ou comportant des équipements d'énergie renouvelable pour les entrepôts, industries et commerce, y compris les parkings couverts de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise, est une bonne chose.

Cet amendement, que je me souviens avoir déjà défendu voilà quelques années, revient régulièrement. Il vise à remédier à des situations bloquantes pour le développement de l'énergie solaire, du fait de la latitude d'interprétation permise par l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme. Par interprétation, certains plans locaux d'urbanisme prévoient l'installation de production d'énergie solaire par intégration au plan de toiture, ce qui suppose le remplacement d'un pan entier entier de l'élément du bâtiment, avec des difficultés en matière d'isolation. Cette approche semble datée, du fait notamment des solutions de surimposition qui se sont désormais imposées, car elles sont à déployer pour les consommateurs, le tarif d'achat majoré des installations intégrées n'ayant plus cours. C'est évidemment moins intrusif sur les structures des bâtiments, moins cher, et cela crée moins de difficultés. Le conditionnement de la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine tels que définis par l'article L. 111-17 du même code permet de prévoir un niveau d'encadrement suffisant

de supprimer la limitation de la dérogation aux seuls cas d'autoconsommation des occupants de l'immeuble. Cette disposition favorisera l'implantation de panneaux photovoltaïques en toiture des immeubles en permettant d'optimiser le dimensionnement de l'installation au regard du potentiel offert par la toiture. La contrainte de l'autoconsommation conduit à limiter le dimensionnement des installations de production d'énergie renouvelable ou à les accompagner d'installations de stockage d'énergie particulièrement onéreuses.

S'ils vont au-delà, ils peuvent être refusés par le permis de construire, alors même que la détermination de la frontière entre les deux est floue. L'amendement n° 336 du Gouvernement vise donc à simplifier l'installation de panneaux solaires et à mettre fin à cette distinction préjudiciable au développement du photovoltaïque. Dorénavant, un permis de construire ne pourra plus s'opposer à l'installation de panneaux solaires, sauf protection du patrimoine historique ou des parcs naturels, même lorsque l'électricité produite est supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer l'autoconsommation. L'adoption des trois amendements identiques n 65 rectifié, rectifié aboutirait, en fait, à l'effet exactement opposé à celui qui est recherché. Ces amendements reviennent à dire que, malgré les règles de protection du patrimoine historique, un permis ne peut pas s'opposer à des dispositifs d'énergie renouvelable. Nous pourrions donc avoir des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments historiques. L'amendement n° 105 rectifié, quant à lui, vise à prévoir quelque chose qui est déjà possible. Aujourd'hui, le droit indique que, malgré les règles du PLU, un permis de construire ne peut s'opposer au photovoltaïque,

ces dispositifs énergétiques, les modalités du calcul des 30 % et enfin certaines dérogations. La méthodologie de calcul est donc simplifiée : désormais, l'obligation s'appliquera à toute création de surface de bâtiment et ombrières de stationnement de plus de 1 000 mètres carrés. Elle pourra être remplie de plusieurs façons : soit en intégrant des dispositifs énergétiques sur la toiture du bâtiment, soit en les intégrant sur les ombrières des parkings, soit sur les deux.

Il n'y a en effet pas lieu de créer un encadrement par le document d'urbanisme du type d'ENR pouvant être réalisée dès lors que l'article L. 151-21 du code de l'urbanisme ne rencontre pas dans sa rédaction actuelle et sur cet aspect de difficulté d'application notoire.

confirment une nouvelle fois que la France est sur la mauvaise voie pour respecter son objectif pour 2020. L'écart entre ce qui est réalisé et l'objectif cible s'est encore agrandi entre 2016 et 2017. Il est donc nécessaire de conforter le développement Le présent amendement vise à préciser et à sécuriser juridiquement les plans locaux d'urbanisme qui souhaiteraient imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements la mise en place d'un système de production d'énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et et la capacité de production attendue. Il s'agit de faciliter la possibilité pour les maires d'imposer l'installation du système de production d'énergie renouvelable. La France prévoyait de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de la consommation finale d'énergie d'ici à 2020. Avec 16,3 % d'énergies renouvelables, la France est le troisième pays dont la part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale brute est la plus éloignée des objectifs.

Or la production d'énergie renouvelable diffère en matière paysagère ou technique selon le type d'énergie retenu. L'article 6 octroie aux maires un outil leur permettant de piloter la cohérence globale des projets énergétiques qu'ils souhaitent voir développés dans certains secteurs en confiant la possibilité au règlement du PLU de définir le type d'énergie renouvelable souhaité dans ces secteurs. La commission y est très attachée.

Cet amendement vise à soutenir, à titre expérimental et dans les territoires couverts par un plan de protection de l'atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement

Quel est l'avis de la commission ? La commission est favorable aux initiatives qui permettent le développement des énergies renouvelables, mais ces amendements reviennent à signer un chèque en blanc sans pouvoir contrôler le rythme ou la cohérence du déploiement de ces dispositifs.